leur permettant de prendre des décisions éclairées et stratégiques, lorsque le moment est venu d'acheter et de fournir ces médicaments au système de santé publique français. Accéder simplement à des informations précises sur le statut de ces brevets est une ressource de grande importance pour que l'État et la société française puissent veiller sur la qualité des brevets délivrés au niveau européen sur les produits thérapeutiques que l'assurance maladie cherche à rendre accessibles aux citoyens français. En 2017, 27 % des brevets délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) ont été révoqués grâce à des oppositions démontrant démontrant l'absence d'application de critères rigoureux ; 42 % ont été maintenus, mais amendés, c'est-à-dire qu'ils ont été modifiés pour mieux correspondre aux critères de brevetabilité. Près de 70 % de ces brevets ont donc été accordés, alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Une telle absence de rigueur de la part de l'OEB devient une menace dès lors qu'elle favorise la création de monopoles sur les biens de santé non soumis à l'exercice du contradictoire, potentiellement octroyés aux dépens des systèmes de santé et des personnes malades.

brevets d'invention en santé prioritaire pour les patientes et les patients sera une importante ressource pour la soutenabilité du régime de l'assurance maladie.

quand la situation sanitaire l'exige, de lever les exclusivités accordées sur certaines licences de produits issus de la recherche publique. Les prix élevés des médicaments innovants sont révélateurs du dysfonctionnement de notre système de recherche et de développement. Financés par des fonds publics, les organismes publics de financement de la recherche, les universités et les instituts de recherche publics ont la responsabilité d'agir dans l'intérêt et au service de la société. C'est d'autant plus vrai lors du transfert de technologies réalisé vers le secteur privé. L'objectif premier de ces institutions doit être de contribuer à la mise en pratique des inventions en santé, tout en respectant le besoin de maximiser l'accessibilité et la faisabilité économique de ces technologies. Il y va de la soutenabilité des systèmes de santé publique. Or les décisions prises lors de la cession de la recherche publique, source majeure dans la constitution de monopoles pharmaceutiques, ne sont pas rendues publiques, ce qui rend impossible tout contrôle et suivi de la part de l'ensemble des parties prenantes du cycle de recherche et de développement. obstacles à l'exercice de la démocratie sanitaire et à la production de politiques publiques rationnelles dans le champ de la recherche biomédicale. Ils sont également l'un des principaux obstacles à la facilitation d'un accès abordable aux technologies de la santé issues de la recherche publique en France et dans le monde. Le présent amendement vise à réduire ces obstacles lorsque la santé de la population est menacée, pour permettre une recherche et un développement soutenables, la délivrance de licences non exclusives étant un moyen dont doit disposer l'État pour atteindre

préalablement à toute modification de ces régimes dérogatoires, en démontrer les limites ou les insuffisances. Par ailleurs, quant à la question plus particulière de l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle issus de la recherche publique, vue de répondre à des besoins d'intérêt général, je souhaite réaffirmer l'importance, pour les établissements, de rester copropriétaires des brevets stratégiques pour la Nation.

à des fins exclusives d'illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche et d'enseignement supérieur publics, à l'exclusion de toute activité à but lucratif.

sans problème. Elle est d'ailleurs autorisée par la directive du 17 mai 2019 et devrait se traduire par une modification de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit déjà plusieurs exceptions, notamment à des fins pédagogiques, au droit exclusif d'un auteur d'autoriser l'exploitation de son oeuvre analyses, courtes citations, représentations, reproductions d'extraits d'oeuvres, fouilles de textes, etc. Ces exceptions ne peuvent s'appliquer aux arts visuels. Outre la fouille de textes, qui ne concernent que les oeuvres écrites, la reproduction partielle d'une oeuvre visuelle constitue une dénaturation de celle-ci et, donc, une violation du droit moral de son auteur.

droit ? Vous le savez, mes chers collègues, et nous le redirons lors de l'examen du projet de loi de finances, les auteurs des arts visuels sont les parents pauvres de la chaîne des droits : pour l'heure, ils n'ont droit à rien. Une licence collective les servirait bien sûr, mais encore faut-il qu'elle soit bien négociée.

Nous ne souhaitons pas du tout refuser la mise en place d'une exception qui servira la recherche, et refuser sa gestion collective en vue de l'attribution d'une juste rémunération au profit des ayants droit, mais il existe un problème de forme : il n'y a aucun débat

l'usage des images pose un problème spécifique qui n'est pas couvert par le droit d'auteur actuel. En effet, il n'est pas possible d'utiliser, par exemple, l'extrait d'un tableau sous peine de violer le droit moral de l'auteur et de perdre en intérêt scientifique dans l'analyse, pas plus qu'il n'est possible de reproduire l'intégralité de l'oeuvre, ce cas n'étant pas couvert par les exceptions au droit d'auteur. L'ordonnance qu'il nous est proposé d'adopter ne crée pas une nouvelle exception aux droits d'auteur, c'est-à-dire un dispositif comme la copie privée, auquel les auteurs ne pourraient pas s'opposer. Cette voie a spécifiquement été écartée au profit de celle de la licence collective étendue, rendue possible par l'article 12 de la directive du 17 avril 2019. Le principe est qu'un ou des organismes de gestion collective jugés représentatifs puissent collecter les revenus et représenter, non seulement leurs affiliés, mais également ceux qui ne sont pas sociétaires. Ma chère collègue, j'entends ce que vous dites, ces auteurs ne sont pas couverts par des OGC et auraient dû se voir proposer une négociation par le ministère concerné.

ce délai étant jugé nécessaire pour mener à bien une concertation approfondie avec les organismes de gestion collective et, donc, avec les auteurs des arts visuels directement, afin de déterminer, en particulier, le montant de la compensation versée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche aux sociétés gestionnaires ou aux auteurs eux-mêmes. Dès lors, les auteurs recevront une rémunération pour de nouveaux usages de leurs oeuvres à la charge du ministère, rémunération négociée- ou pas -par leurs représentants, régime dont ils peuvent choisir de se retirer à tout moment. L'équilibre atteint me paraît satisfaisant et l'ordonnance justifiée par l'absence actuelle de licence collective dans notre droit. Je suis défavorable à cet amendement de suppression.

Mon cher collègue, le crédit d'impôt recherche suscite des débats récurrents, à la fois sur son ampleur, plus de 6 milliards d'euros, et sur la possibilité de mieux le cibler, par exemple en y adjoignant des objectifs environnementaux ou en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le cas présent, les auteurs sont plus respectueux de sa vocation, mais je ne suis pas persuadée de l'applicabilité de cette mesure. Tout d'abord, tous les travaux de recherche n'ont pas vocation à donner lieu à publication, surtout quand cette recherche est appliquée. Ensuite, je crois que nous aboutirions à une véritable usine à gaz, qui permettrait à l'administration de réclamer un remboursement du crédit d'impôt recherche. Bref, un cauchemar administratif de plus ! Je vous invite cependant à rouvrir ce riche débat lors de l'examen du projet de loi de finances. Avis défavorable.

il précise que c'est bien l'ensemble des activités qui contribuent à l'ensemble des missions prises en compte pour l'évaluation et, partant de là, pour la progression des carrières. Je suis très attachée à cet article, et c'est pourquoi je suis défavorable

je crois qu'il est important de rappeler que les deux premières missions des enseignants-chercheurs sont bien sûr de chercher et d'enseigner. Ils manquent déjà de temps pour les mener à bien sereinement et on leur en ajoute sans cesse, sans compter le temps qu'ils doivent employer à répondre à des appels à projets, dont dépend de plus en plus le financement de leurs recherches. Même si l'intention est louable, il n'est pas certain qu'il soit raisonnable de demander à ces enseignants-chercheurs de se disperser encore davantage. L'ajout d'une nouvelle tâche n'est pas réaliste.

Je comprends bien que l'introduction de cet article dans le projet de loi a été motivée par l'actualité : la crise sanitaire que nous traversons a entraîné une accélération de la circulation de fausses informations scientifiques, et je salue le fait que cela nous donne l'occasion d'en parler : c'est important. Mais une autre actualité m'incite à refuser que notre société se décharge d'une mission de plus sur ces enseignants sans se demander s'il est techniquement possible pour eux de la mener à bien. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ? Madame Monier, je serai d'autant plus défavorable à votre amendement

En effet, le CSA a déjà un rôle dans la lutte contre les de manière générale ; il a donc une vocation naturelle à intervenir aussi contre les scientifiques. Pour ce faire, nous proposons que le CSA fasse un bilan de l'activité du réseau Science et médias » dans son rapport annuel, plutôt que de créer, comme nous en avons trop souvent l'habitude dans notre pays, une nouvelle entité indépendante de toute autre structure. Ainsi, le CSA superviserait le réseau « Science et médias Mon cher collègue, le centre « Science et médias » fait partie des projets dont il est fait mention à l'alinéa 212 du rapport annexé. Il aurait pour mission d'assurer une bonne diffusion de la culture et des informations scientifiques en mettant en relation journalistes et chercheurs. Le lien avec le CSA n'est en réalité pas évident,

-par François Germinet, président de l'université de Paris-Cergy, en novembre 2015, sur la promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce rapport soulignait, si besoin était, le potentiel de développement des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dans le marché de la formation continue. Il préconisait, par exemple, la création de sociétés d'accélération de la formation continue sur le modèle des sociétés d'accélération du transfert de technologies.

L'élection à la majorité absolue des membres du conseil d'administration peut conduire à des situations de blocage. Il est nécessaire d'imposer un mode de scrutin qui permette une élection rapide des présidents d'université. Cette nécessité ne doit pas remettre en cause l'esprit du scrutin, celui de la recherche du consensus au sein des différents corps représentés. L'élection au scrutin préférentiel alternatif à un tour paraît de ce point de vue la plus adaptée, car elle garantit l'élection rapide d'un président consensuel, avec un soutien large au sein du conseil d'administration.

Enfin, les contentieux récents imposent de clarifier les règles d'éligibilité aux fonctions de président d'université. Notre proposition s'inscrit dans la logique des travaux préparatoires de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2017, en permettant une ouverture large du champ des catégories de personnels éligibles à la charge de président d'université. J'en profite pour vous informer que nous retirons d'ores et déjà les amendements n 13 14 et 15.

au sein des comités territoriaux de recherche en santé, une politique de valorisation de la recherche publique responsable. À travers celle-ci, il s'agirait de faciliter la transparence et la traçabilité des innovations financées par des fonds publics et de rendre ainsi les médicaments, par exemple, plus accessibles et soutenables en termes de coûts. Dans cet esprit, nous proposons que le président d'université présente chaque année au conseil d'administration, en collaboration avec les comités territoriaux, un rapport sur la politique de valorisation de la recherche publique responsable. En tant que piliers du système de recherche français,

Les universités hébergent une part non négligeable de la recherche publique biomédicale en France. En tant qu'organismes financés sur des fonds publics, elles ont la responsabilité d'agir dans l'intérêt et au profit du public. Dès lors, toute technologie de santé issue de la recherche financée par des fonds publics et ayant le potentiel de devenir un médicament, un vaccin ou un dispositif médical devrait être transférée selon une stratégie concrète et transparente, visant à permettre un accès équitable et à mettre à la disposition des patients des versions abordables de cette technologie. Le présent amendement vise donc à ancrer la responsabilité sociale de l'établissement en termes de recherche, et ce au plus haut niveau de gouvernance. Les modalités de la collaboration entre l'université et la société d'accélération du transfert de technologies dont elle dépend devront être fixées par décret.

relève d'acteurs extrêmement variés : les centres hospitaliers- lesquels ne sont pas forcément universitaires -, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les organismes de recherche, éventuellement d'autres universités.

Nous avons voté plusieurs amendements forts en faveur des libertés académiques, au titre desquelles le président d'une université ne représente pas l'État

ici, de rien d'autre que de garantir, dans certaines circonstances très exceptionnelles- je dis bien très exceptionnelles -, la bonne marche de l'université et la qualité des diplômes. Si, comme vous le savez, les présidents d'université sont les garants, dans la loi, de l'ordre public et de l'organisation matérielle des examens, « loi Fioraso », a transmis la compétence de fond sur les modalités des examens aux commissions de la formation et de la vie universitaire. Or, à quelques reprises, ces commissions ont pris des décisions à la légalité douteuse, par exemple l'attribution de la moyenne à l'ensemble des étudiants. Que peut alors faire le président ? Il ne dispose que de recours très limités, ce qui le met évidemment en porte-à-faux. Il doit demander au recteur de saisir le tribunal administratif, ou au ministre d'utiliser, lorsque les circonstances l'exigent, toutes les mesures nécessaires.

Or l'organisation et la gouvernance de l'université des Antilles ne lui ont pas permis de parvenir à un fonctionnement satisfaisant de ses instances, en dépit d'une structuration décentralisée des établissements en pôles universitaires, autant dans la région de Guadeloupe que dans celle de Martinique. Cet amendement vise donc à inscrire le principe selon lequel la désignation du président de l'université et de ses deux vice-présidents fera l'objet d'un seul et même vote par le conseil d'administration

le cas d'un vice-président, le président d'université proposera au conseil administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Cet amendement entrerait en vigueur lors de la désignation du prochain président de l'université des Antilles.

2015 ! À l'époque, il fallait absolument éviter une partition. La Guyane étant déjà partie, il fallait tenir le pôle de Martinique et le pôle de Guadeloupe en une seule et même université. Il y avait cette exigence politique-

Avec cet amendement, nous proposons qu'il ne soit possible de donner mandat qu'à des organismes publics. Ces six institutions incarnent l'excellence française dans leur domaine respectif ; elles font partie de notre patrimoine intellectuel commun. Il est de notre devoir, nous en sommes convaincus, de nous assurer que leur gestion financière reste dans le domaine public.

pour l'État, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, les collectivités locales et leurs établissements publics. Je mets aux voix

permettant aux chefs d'établissement de bien garder autorité sur les personnels d'enseignement et de recherche, de s'assurer que ces agents ne négligent pas leur activité principale au profit des activités autorisées dans le cadre du cumul.

Cet encadrement pourrait effectivement se révéler utile dans certains cas : il paraît assez légitime, si l'activité annexe se fait au détriment de l'activité principale, que le chef d'établissement puisse y mettre un terme ou la réduire.

il n'est plus temps de leur permettre de trouver un stage. Ce dont ils ont besoin, c'est de trouver un travail, à travers un contrat stable, pour pouvoir s'investir pleinement dans leur nouveau projet de recherche. Nous devons être en mesure d'offrir à nos doctorantes et à nos doctorants de véritables perspectives d'embauche après leur diplôme.

permettant à des chercheurs doctorants de mettre leur expérience et leurs compétences à disposition d'une administration ou d'une entreprise : ce sont eux qu'il faut encourager.

Nous nous situons ici dans le cas où un doctorant, hors de son champ de compétences, souhaiterait effectuer un stage dans un autre univers. Cela ne me paraît en rien incompatible avec une carrière universitaire et cela repose sur le libre choix du doctorant, d'autant plus que la période de stage ne sera pas décomptée de sa période de thèse. L'avis est défavorable. n° 121 rectifié m'apparaît un peu trop large, puisqu'il vise l'ensemble des césures effectuées sous forme de stage, y compris celles qui ne sont pas faites par les doctorants. De plus, il ne me paraît pas pertinent de compter, dans la validation de la formation doctorale, des stages qui pourraient n'avoir qu'un lien réduit avec cette formation. Ce serait même dangereux ! L'avis

vise à donner les moyens législatifs aux autorités compétentes- autorités ministérielles ou établissements -pour mettre en oeuvre des dispositifs assurant un recrutement diversifié des étudiants. C'est une promesse de la République que d'offrir à tous ses enfants la possibilité d'accéder à toutes les filières d'enseignement, y compris celles qui sont parfois considérées, par certains, comme les plus prestigieuses. Il appartiendra donc aux autorités compétentes de fixer, par voie réglementaire pour les administrations ou par les instances de l'établissement lorsque le décret statutaire leur en donne la compétence, les modalités permettant d'atteindre cette diversité parmi les élèves.

Je rappelle que les licences professionnelles étaient initialement destinées à des élèves pouvant avoir eu un parcours chaotique. L'évolution de ces formations les a rendues sélectives et elles sont sans cesse davantage dévoyées de leur objet premier : rendre les études accessibles à toutes et à tous, notamment aux bacheliers techniques, voire professionnels.

et seuls ceux qui ont obtenu une bonne mention y sont généralement acceptés. Que reste-t-il pour les élèves issus de baccalauréats techniques et pour les élèves titulaires d'un « bac pro » ? Nous sommes entrés depuis des années dans une spirale infernale, que nous allons accentuer

en formation complète de niveau bac+3. Tel n'était pas le cas avant cette date, où les étudiants de STS ou de brevet de technicien supérieur- BTS -rejoignaient en troisième année la licence professionnelle à l'université ou en IUT. Avec cet arrêté, la licence professionnelle se trouve dans une situation paradoxale : ou bien elle est préparée dès la première année après le baccalauréat dans un IUT et elle demeure sélective, ou elle est préparée au même stade dans une université et elle ne peut plus l'être, car l'université ne pratique pas, sauf mention spécifique, de sélection à l'entrée. Les alinéas que les auteurs de l'amendement proposent de supprimer visent donc à clarifier le régime des licences professionnelles préparées à l'université, en les rendant sélectives. Cela ne modifie pas la situation actuelle- cette licence est déjà sélective -, mais met en cohérence le niveau législatif avec l'arrêté réformant cette formation.

portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat pourront signaler dans leur dossier de saisine leur situation particulière. Cet amendement a pour objet d'assurer que le traitement de ces informations fournies par les étudiants suit une seule et même procédure et que chacun des étudiants en situation de handicap handicap dispose du même niveau d'accompagnement. En outre, le dispositif actuel ne permettant pas de proposer à tous les étudiants qui saisissent le recteur une poursuite d'études en première année de master en tout point conforme à leur projet, cet amendement a pour objet de créer un nouveau droit pour les étudiants en situation de handicap bénéficieront d'un droit de saisine particulier du recteur de la région académique afin de demander le réexamen de leur situation et d'obtenir, par décision dudit recteur, une affectation dans une formation du deuxième cycle compatible avec leurs besoins.

Mme Sylvie Robert. Cet article reprend, pour les généraliser sans limitation dans le temps, les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Il permet de déroger aux dispositions légales et réglementaires fixant les modalités d'accès à toutes les formations d'enseignement supérieur dispensées par l'ensemble des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes ouvrant à toutes les formations d'enseignement supérieur, « y compris le bac », si l'autorité compétente estime qu'une « situation d'urgence » le justifie. Quant Quant au périmètre des dérogations, il est très large : y figurent la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d'organisation des épreuves aux examens et concours, qui pourront notamment s'effectuer de manière dématérialisée. L'absence de définition de la notion de « conséquences de situation d'urgence », élément potentiellement déclencheur de ces adaptations au droit commun de l'organisation des épreuves et de délivrance des diplômes, est extrêmement préoccupante et n'est pas de nature à nous rassurer.

sans contours précis ni limitation dans le temps. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, qui entame le principe d'égalité de traitement des candidats aux examens et concours. Malgré les affirmations de principe, ce dispositif laisse la place à l'arbitraire. Surtout, il pourrait porter un coup de canif supplémentaire au caractère national des diplômes et des formations

des fins scientifiques. Actuellement, dans ce cas de figure, les promoteurs de recherches doivent obtenir une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, ou l'avis favorable d'un comité de protection des personnes (CPP). Ils doivent ensuite adresser une demande d'autorisation d'importation ou d'exportation au ministère.

à Mme Claudine Lepage. Nous sommes opposés à la ratification de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette ordonnance permet trois types d'organisation.

par des établissements liés par une convention ; une convention détermine alors les compétences exercées en commun par les établissements participant au rapprochement, leurs modalités d'exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination. Enfin, un établissement expérimental- c'est le dispositif le plus intégrateur -peut regrouper ou fusionner des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Les établissements regroupés dans l'établissement public expérimental n'en peuvent pas moins conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l'établissement public expérimental. Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul établissement public expérimental. L'application de cette ordonnance va donc avoir un impact très concret dans les territoires. Elle va entraîner une grande confusion dans le paysage universitaire territorial.

S'agissant des expérimentations organisées sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, le Conseil d'État rappelle que la dérogation au principe d'égalité devant la loi n'est possible que pour une expérimentation ayant un objet limité et pour une durée qui, tout en étant suffisante, doit être strictement nécessaire et que l'objet de ces expérimentations ne peut, par suite, consister en la création de dispositifs dérogatoires permanents

que seules les Comue préexistantes peuvent faire évoluer leur statut. C'est cette ambiguïté que j'ai souhaité lever. En réalité, deux hypothèses se font jour. La première est celle d'une Comue préexistante souhaitant devenir une Comue expérimentale.

Cela n'est possible que si le périmètre de la Comue expérimentale est strictement le même que celui de la Comue préexistante. La seconde est celle d'une Comue expérimentale créée. Cette création entre directement dans le champ de l'expérimentation

transformations dont il s'agit sont soumises aux instances des établissements membres

de rendus d'avis sur les biotechnologies, sans compter de nombreuses modifications du code de l'éducation. Je me félicite que l'examen du projet de loi en commission ait déjà permis de retirer du champ de l'ordonnance certains de ces sujets,

Il n'est pas concevable de légiférer sur ces questions dans la discrétion des cabinets ministériels, la Nation et ses représentants doivent s'en saisir ; c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

de risque nul ou négligeable d'organismes génétiquement modifiés. Simplifier, mais de quelle manière ? Les manipulations en milieu confiné sont des opérations durant lesquelles les OGM sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de manière à limiter leurs contacts avec l'environnement et la population.

dans les mains du seul Gouvernement ; c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet alinéa. Le sujet traité par cette habilitation est très technique. Je me lance ! La procédure actuelle concernant l'utilisation confinée d'OGM à risque nul ou négligeable est particulièrement complexe et va au-delà des exigences de la directive du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés. En particulier, chaque usage doit faire l'objet d'une déclaration transmise au Haut Conseil des biotechnologies (HCB), ce qui constitue une contrainte administrative très lourde. Le projet d'ordonnance viserait donc à aligner strictement la procédure française sur les standards européens, avec mise à disposition Il me semble donc que, dans le cadre de la lutte menée par le Sénat contre les surtranspositions, cette ordonnance pourrait être utile. L'avis est donc défavorable. Quel est

à des contraintes réglementaires plus lourdes que celles qui s'appliquent à leurs collègues européens. Il s'agit également de permettre aux agents chargés du contrôle des utilisations d'OGM de se concentrer sur les utilisations relevant des classes de confinement de deux

mesures techniques ce projet de loi. Le sens des évolutions que nous nous proposons d'adopter par voie d'ordonnance, si vous nous y autorisez, est clairement annoncé. C'est pourquoi l'avis du Gouvernement

Le Haut Conseil des biotechnologies est chargé d'éclairer le Gouvernement sur les questions relatives à l'usage des biotechnologies et d'émettre des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter, par exemple, l'utilisation confinée ou la dissémination d'OGM. Cette structure a montré des difficultés importantes à fonctionner depuis sa création, et notamment à conduire sereinement les débats entre parties prenantes. Des vagues de démissions ont, à plusieurs reprises, entraîné le blocage de son comité économique, éthique et social et ont fragilisé son comité scientifique. Pour consolider et pérenniser les fonctions d'évaluation indispensables à l'éclairage de la décision publique sur les biotechnologies, il est nécessaire de s'assurer d'une évaluation des risques rigoureuse, indépendante et de qualité, de confier à des experts une analyse économique des bénéfices sociaux des biotechnologies amenées à être développées, d'aborder avec compétence les questions éthiques et de donner sa place à un vrai débat public dans le cadre duquel toutes les composantes de la société pourraient s'exprimer. Le Gouvernement envisage donc de transférer les missions actuelles du Haut Conseil des biotechnologies à différentes instances déjà existantes, robustes et reconnues, qui seront capables d'intégrer ces nouvelles missions dans leur fonctionnement. C'est le cas de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui se verra confier la mission d'évaluation des risques environnementaux liés à la dissémination d'OGM. Cette agence possède une forte expertise dans les domaines environnementaux, sanitaires et agronomiques, et sa pratique de l'évaluation des risques est confirmée et reconnue, puisqu'elle délivre déjà des avis sur les risques sanitaires liés à cette même dissémination d'OGM. L'Anses se verra également confier la mission d'analyse socio-économique et mettra en place, à ce titre, un nouveau comité d'experts spécialisés dans ce domaine. plus, le Gouvernement envisage de transférer au ministère chargé de la recherche la mission d'évaluation des dossiers de demande d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, en plus des missions de délivrance de ces autorisations et de contrôle qu'il exerce déjà. Enfin, le Gouvernement examine la possibilité de faire du Conseil économique social et environnemental le siège du débat public sur les biotechnologies et de confier au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé l'examen des questions éthiques qui leur sont relatives. L'objectif de cet amendement est de faciliter cette réorganisation pour assurer la nécessaire continuité de l'expertise sur les biotechnologies ; le recours à une ordonnance est lié à la technicité de ce sujet

? Cet amendement tend à revenir sur un vote clair exprimé en commission sur un amendement de la commission des affaires économiques. Il me paraît important de bien marquer l'opposition du Sénat à la multiplication des ordonnances. L'avis est donc défavorable.

amendement ne permet pas de savoir comment seront traités les sujets plus précis, comme la recherche sur les médicaments de thérapie génique ou les applications en matière de défense nationale.

l'habilitation. Ces explications sont bienvenues, mais notre position de principe reste, sur les sujets qui ne sont pas purement techniques, la suppression.

lequel autorise le Gouvernement à modifier le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l'utilisation des semences de variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH) et des produits qui en sont issus. issus. Ces variétés ont été rendues tolérantes aux herbicides par des techniques conventionnelles, par la sélection traditionnelle ou transgénique. Ces semences posent un certain nombre de problèmes, notamment le développement de résistance des adventices, c'est-à-dire des mauvaises herbes, aux herbicides et l'augmentation de l'utilisation d'herbicides par rapport à des cultures classiques, entraînant,, la contamination des milieux. Encore une fois, ce débat ne doit pas être pris à la légère. Personne ne s'étonnera de voir des écologistes se saisir de ce dossier,

de la commission ? Là encore, le sujet est technique, et la ministre pourra certainement compléter mon propos. L'avis de l'Anses du 26 novembre 2019 juge nécessaire l'instauration d'un suivi des variétés rendues tolérantes aux herbicides. Par un arrêt du 7 février 2020, le Conseil d'État a estimé que ce suivi était nécessaire. L'ordonnance a pour objet de modifier le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de le rendre possible.

des mesures relevant du domaine de la loi concernant l'enseignement supérieur privé. Il vise à mieux expliciter les finalités de cette habilitation concernant l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur et la délivrance des diplômes. En ce qui concerne le régime d'ouverture, dans un souci de clarification et de simplification, il s'inspirera du régime prévu par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

en vigueur : la reconnaissance d'établissements d'enseignement supérieur technique, lesquels, une fois qu'ils sont reconnus, ne demandent plus rien à personne, si je puis dire,

de manière à être en mesure de vérifier les titres et travaux des personnes qui enseignent dans ces établissements, mais aussi de garantir la meilleure information possible aux parents, lorsque ceux-ci inscrivent leurs enfants

Je tente ma chance pour la troisième fois ... Le présent amendement a pour objet de rétablir l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance sollicitée par le Gouvernement en matière spatiale. Quel est

au ministère des armées d'opérer des dispositifs spatiaux sans intermédiaire et de revoir le régime de déclaration préalable à l'utilisation de données spatiales afin de rendre crédibles les stratégies spatiales de défense. l'habilitation permet d'aller beaucoup plus loin et de procéder à une refonte globale de la loi sur les opérations spatiales, qui mérite un vrai débat, surtout sur des sujets aussi importants que l'encadrement des mégaconstellations et des activités industrielles dans l'espace. Un groupe de travail a formulé quarante-sept propositions sur quatorze thématiques, dont nous n'avons pas connaissance en l'état.

au secteur privé. S'il faut former davantage de vétérinaires, faisons le choix d'ouvrir une nouvelle école publique ou ouvrons de nouvelles places dans les écoles existantes en leur donnant les moyens de le faire. Autoriser la création d'écoles vétérinaires privées aurait un coût important, dont le financement se ferait sans doute au détriment des établissements publics ; pourquoi ne pas plutôt faire le choix d'utiliser les sommes correspondantes pour aider nos écoles de vétérinaires publiques à augmenter leur capacité ? Peut-être pourrions-nous en discuter le mois prochain, lors de l'examen du projet de loi de finances ? Quel est l'avis de la commission ? Cet article a été introduit en commission par la présidente Sophie Primas et le président François Patriat ; il me semble qu'il a été longuement concerté avec les professionnels

Vous êtes bien taquin, monsieur le président ! Madame la ministre, permettez au vétérinaire présent dans cette assemblée de donner son sentiment. Notre profession vit un véritable paradoxe

en ville, paradoxalement, à l'inverse de ce que tout le monde croit. Les vétérinaires praticiens libéraux ont beaucoup de mal à recruter des salariés pour faire le travail.

de soutenir financièrement ce type d'exercice me paraît beaucoup plus adaptée qu'une éventuelle augmentation du nombre de places au concours- ou d'ailleurs que la création de places dans une école vétérinaire privée à but non lucratif.

à diminuer la capacité de recherche dans ce domaine et à précariser l'offre de formation publique. Les moyens qui seraient transférés à cette école vétérinaire privée doivent rester destinés à l'enseignement vétérinaire public, pour lui permettre d'augmenter ses capacités d'accueil. d'accueil. Fragiliser une nouvelle fois le service public de recherche et de formation ne paraît pas judicieux, à l'heure où l'on a besoin d'une recherche vétérinaire forte pour adapter l'agriculture aux défis environnementaux et de santé publique, qui sont liés notamment à l'antibiorésistance et à la nécessaire amélioration du bien-être animal en élevage.

faut-il que toutes ces techniques soient bien connues par celles et ceux qui ont à travailler dans le milieu de l'expérimentation ! Par ailleurs, la directive européenne 2010-63, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, représente, selon ses propres termes, « une étape importante vers la réalisation de l'objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que cela sera possible sur un plan scientifique ». Dans ce cadre, a pour objet de faire connaître toutes les techniques de substitution aux étudiants des filières biomédicales, qui auront, à un moment quelconque, à se mesurer aux questions expérimentales, afin de diminuer le recours aux animaux vivants pour ces expérimentations. J'ajoute que la fiabilité des nouvelles techniques est considérablement supérieure à celle de l'expérimentation animale

Dans le même temps, en Grande-Bretagne, on en utilisait vingt fois moins. Si nos collègues d'outre-Manche étaient beaucoup moins bien formés que les étudiants français, cela se saurait

on peut avoir recours à des méthodes de substitution tout à fait suffisantes, telles que les vidéos en 3D, les mannequins et des outils de simulation, d'ailleurs très appréciés des enseignants et des étudiants.

comme cela s'est produit avec les cosmétiques : depuis 2009, ceux-ci ne peuvent être commercialisés dans l'Union européenne que si ni les composants ni le produit fini n'ont été testés sur des animaux. L'industrie cosmétique était, à l'époque, opposée à cette réglementation

encore jeune, puisqu'elle a été créée sous cette forme en 2015, sur l'initiative du ministère de l'agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt. visait à améliorer la coopération entre l'enseignement supérieur et la recherche agronomique, vétérinaire et forestière, afin d'acquérir une meilleure renommée internationale dans ces domaines et d'être en mesure de former les chercheurs et chercheuses qui inventeront de nouvelles solutions pour réussir la transition agroécologique. En particulier, l'institut devait permettre une meilleure coordination entre les différents établissements, pour qu'ils mènent des stratégies communes et élaborent des projets en commun. La recherche agronomique, vétérinaire et forestière est indispensable,

Les promesses se sont transformées en une reconduction du croît budgétaire famélique que votre ministère connaît depuis 2017. La correction apportée par le Sénat à cette programmation budgétaire est quelque peu salvatrice. J'incite vivement notre rapporteure à la défendre jusqu'au bout en commission mixte paritaire. De cette loi de programmation budgétaire sans budget, il restera des dispositions qui poursuivent et amplifient le processus ininterrompu de dislocation du service public. C'est un paradoxe, car j'avais cru comprendre de nos débats vos velléités de refuser le modèle anglo-saxon, dont nous n'avons pas assez dit qu'il est profondément en crise. Si notre pays accepte l'idée que la connaissance est une marchandise et que la concurrence sans limite doit être son mode de régulation, alors nous sommes perdus Car jamais votre ministère ne pourra doter nos établissements de capacités financières suffisantes pour lutter dans cette compétition. Je reste persuadé que le service public constitue un cadre plus propice à la recherche, car il donne aux chercheurs une stabilité qui favorise la prise de risque et la recherche de longue haleine ; au même moment, il garantit à l'État l'indépendance de ses chercheurs au service de l'intérêt général. Nos chercheurs attendaient de nous de la confiance : je ne comprends pas comment nous avons pu passer d'une déclaration faisant des libertés académiques les conditions de l'exercice et de l'excellence de la recherche à une formule qu'ils perçoivent comme une atteinte à ces mêmes libertés. De la même façon, pourquoi affaiblir le Conseil national des universités dans son rôle de garant de la valeur nationale des grades universitaires ? Il serait opportun de corriger ces deux points en commission mixte paritaire. Pour conclure, je reprendrai une formule qui convient malheureusement bien à une communauté dans laquelle la moitié des salariés sont précaires

ce sous-financement n'est pas le résultat d'une calamité naturelle : ce n'est pas le puceron vert qui a grignoté le budget de la recherche année après année ; c'est bien la logique d'austérité qui a conduit la recherche française dans une situation qui nous oblige aujourd'hui à rattraper les erreurs passées.

Sur les budgets que vous aurez à défendre, madame la ministre, l'effort reste largement insuffisant. Le courage du verbe, mais l'absence d'actes concrets : pour l'écologie comme pour le reste, c'est encore et toujours pareil ! En revanche, pour précariser ou affaiblir les statuts des chercheurs, on remarque une certaine gourmandise de votre part : vous n'alliez tout de même pas vous priver d'affaiblir une nouvelle fois le CDI ou les statuts de la fonction publique. Une programmation budgétaire insuffisante, une précarisation des parcours professionnels, l'organisation de la compétition entre universités et des annonces antiécologistes : tous ces éléments sont constitutifs d'un texte au mieux inefficace, au pire dangereux pour le monde de la recherche- un texte qui ne mérite pas l'appellation de programmation. Votre texte se fait contre la communauté universitaire : les réseaux d'enseignants-chercheurs, la société civile et les associations nous alertent depuis des semaines et ont été atterrés par certains de nos débats au Sénat. En réduisant la programmation budgétaire de dix à sept ans, le Sénat avait pourtant remis un peu de cohérence entre les ambitions et la réalité. Mais les amendements votés ces derniers jours ont aussi conduit à des reculs supplémentaires qui suscitent de très vives inquiétudes, sur les libertés académiques académiques comme sur le mode de recrutement du corps enseignant, dont le processus a été radicalement changé. Nous voterons donc contre ce texte, qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu financier et qui prolonge une vision de l'université en compétition permanente, conduisant à son affaiblissement. La

Nous avons eu de beaux débats sur les libertés académiques- ceux qui veulent affoler en seront largement pour leurs frais -, ... Tout à fait ! ... sur l'intégrité scientifique, sur l'évaluation des établissements, sur la diversification nécessaire des contrats pour permettre à de jeunes talents de trouver de trouver leur place. Nous avons eu des débats récurrents sur les crédits d'impôt et leur utilité, cher Pierre Ouzoulias. Nous avons un point de divergence sur l'intensité de l'effort,

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un prix Nobel de chimie attribué à une brillante chercheuse française expatriée en Allemagne, n'est-ce pas là le symbole de ce que nous devons éviter : la perte d'attractivité de la France en tant que grande nation scientifique ? Pour éviter le décrochage de notre pays dans le domaine de la recherche, le projet de loi fixe un objectif ambitieux en termes de moyens budgétaires. Le groupe du RDSE partage l'avis de la commission, qui a ramené le cap de la programmation à 2027. Il y a urgence à agir, la compétition mondiale étant de plus en plus aiguë.

Mes chers collègues, la pandémie de covid-19 nous rappelle hélas dramatiquement combien la recherche est un défi permanent pour le bien de l'humanité. Enfin, d'un point de vue davantage philosophique, philosophique, la recherche, lorsqu'elle interroge la science, est une façon de mieux connaître le monde. À l'heure où un certain obscurantisme menace tragiquement notre société, notre responsabilité est d'encourager le progrès à tous les niveaux. Par conséquent, le groupe du RDSE votera pour ce projet de loi. La parole vote. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte était très attendu par la communauté scientifique, qui exprime depuis longtemps le besoin d'une véritable revalorisation du financement de la recherche.

nous regrettons d'avoir été contraints d'examiner ce texte en procédure accélérée et dans l'urgence, au lieu de prendre le temps de construire collectivement un projet à long terme pour l'excellence de la recherche française, car, ce soir, le résultat n'est pas satisfaisant.

Pour leur donner réellement la possibilité de prendre le temps, ce temps si indispensable aux grandes découvertes, la recette est simple : il faut des financements pérennes et des contrats stables et sécurisants. Le texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer ne repose ni sur l'un ni sur l'autre. Plutôt que de privilégier le financement de la recherche fondamentale dans tous les domaines, il fait la part belle aux financements par appel à projets, l'ANR, alors que nous savons que nos chercheurs et nos chercheuses s'usent dans les procédures

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avions l'occasion de bâtir un avenir radieux pour la recherche française, et de sortir de cet hémicycle en étant fiers d'être parvenus à renforcer notre service public de la recherche, pour qu'il soit prêt à faire rayonner la France sur la scène scientifique internationale et que nos plus brillants esprits soient ceux qui inventeront le socle d'une transition écologique et sociale heureuse. Il n'en est rien ! Notre collègue Sylvie Robert nous avait indiqué que nous appelions de nos voeux un miracle. Force est de constater qu'il n'a pas eu lieu. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc contre ce texte, qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. La parole est

Ce projet de loi de programmation est l'objet de vives critiques d'une partie de la communauté des chercheurs. Nous devons faire la part des choses entre l'expression des craintes de personnes ayant une rente de situation dans notre pays et des revendications tout à fait légitimes,

juniors. C'est un travail constructif, qui va dans le sens d'une bonne recherche. Ce texte qui prévoit d'allouer 25 milliards d'euros supplémentaires sur sept ans au financement de la recherche, replace la science, l'innovation et la volonté de comprendre et d'entreprendre au coeur de notre société. Il favorise le recrutement de jeunes chercheurs hors norme, ces moutons à cinq pattes qui passent souvent entre les mailles des concours habituels et des grilles de lecture classiques

le rééquilibrage entre des nouveaux contrats, dont j'estime qu'ils doivent trouver leur place dans certains systèmes, tout en ménageant un équilibre par rapport aux carrières et aux contrats déjà existants,

Le scrutin est ouvert.

donc une forme d'humilité. Au nom de l'ensemble des personnels de la recherche, je tiens à remercier le Sénat de ce vote.

jamais les libertés académiques ne pourront pâtir du respect des valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et le refus de toutes les discriminations. J'informe le Sénat les discriminations. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental et sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ne sont pas parvenues à l'adoption d'un texte commun.